pour des opérations complexes ou dans des terrains difficiles, et cela arrive plus qu'on ne le pense dans les reliefs chahutés des îles.

Or les articles 199 C et 217 prévoient que, lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. Ainsi, entre le moment de la clôture de la souscription et l'achèvement de l'immeuble, quatre ans peuvent s'écouler, ce qui apparaît comme une durée suffisante. Un allongement de cette durée pourrait entraîner un réel dévoiement de l'avantage fiscal. La commission a estimé qu'il s'agissait d'un délai suffisant et a émis un avis défavorable.

de l'article 199 C pour les particuliers et pour celles et ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu jusqu'en 2025, avec des conditions supplémentaires de contrôle, notamment d'agrément des

Des gouvernements sont passés et ont abîmé cette stabilité fiscale. Chaque année, en loi de finances, on peut remettre en cause les dispositifs. La preuve, nous le vivons encore cette année.

à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, sauf dans les DROM, où l'on verrait ultérieurement. Il ne s'agit pas d'une histoire de coût, mais il convient de donner de la stabilité pour qu'un investisseur puisse être rassuré.

au mois de juillet 2018. La baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui passera de 33 % en 2018 à 25 % en 2022, va avoir un impact négatif sur les schémas de défiscalisation à l'impôt sur les sociétés. Elle va réduire de 10 à 13 points l'attractivité de ces schémas, du fait de la réduction de la base éligible, elle-même liée au taux d'impôt sur les sociétés. Je propose par cet amendement de maintenir au même niveau l'avantage fiscal par un coefficient de révision, ce qui permettra d'annuler l'effet négatif de la baisse de l'IS. Cet amendement a déjà été débattu à l'Assemblée nationale. Je souhaite avoir confirmation que ce sujet d'importance pour les collectivités françaises du Pacifique sera bien pris en compte.

Le présent amendement a pour objectif de donner aux représentants de l'État dans les départements d'outre-mer la possibilité d'agréer une opération de construction de logements intermédiaires au bénéfice du taux réduit de TVA, sans que la condition du minimum de 25 de surface de logements sociaux ait à s'appliquer. Ces opérations sont destinées à la location à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 du code Il aligne, pour les départements d'outre-mer, où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd'hui un véritable enjeu, les conditions d'éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui font l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi du loi du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

la procédure d'élaboration de la loi fiscale, car on voit bien que notre procédure est insatisfaisante, incomplète et insuffisamment rigoureuse. Nous devons prendre le temps de garantir la robustesse juridique des dispositifs votés. » Quel auteur

parlons. Sur la méthode, ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur général, j'aurais pu le dire au cours des dix années précédentes, pour avoir siégé à l'Assemblée nationale et avoir regretté maintes fois que des amendements du gouvernement soient présentés tardivement. Je tiens cependant à indiquer, au-delà de ce constat et des excuses que je présente à votre assemblée, que le principal des modifications et du dispositif est contenu dans les articles du projet de loi de finances initial, que les amendements que nous avons déposés tardivement sont des amendements d'ajustement visant justement à sécuriser le dispositif pour les entreprises, nés de travaux de concertation menés jusqu'à la dernière minute. Je ne suis pas convaincu, monsieur le rapporteur général, de pouvoir vous donner ma parole et celle du Gouvernement que plus jamais, ô grand jamais, cela ne se reproduira, car nous savons l'un et l'autre

12 vise à mettre le régime de l'intégration fiscale en conformité avec le droit européen, tout en garantissant « l'attractivité »- le grand mot à la mode ces temps-ci -du dispositif. Pour ce faire, il est proposé de réduire le taux de quote-part des frais et charges de 12 % à 5 % pour l'ensemble des entreprises. Or ce dispositif, qui exonère largement les groupes fiscalement intégrés d'imposition sur les plus-values de cessions intragroupes de titres de participation, n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse quant à son impact sur les finances publiques. publiques. Une simulation aurait été réalisée chiffrant la présente mesure à 330 millions d'euros par an, hors opérations exceptionnelles. Évidemment, ce sont essentiellement les grandes entreprises, les transnationales et les holdings possédant de multiples filiales qui sont concernées par ce dispositif. Ainsi, cette mise en conformité avec le droit européen n'entraînera pas de coût pour ces entreprises, puisqu'il est proposé d'élargir la « niche Copé ». Or cette niche enfle année après année.

Nous avons précédemment débattu de l'opportunité de supprimer de très nombreuses niches fiscales dont le coût était faible et qui bénéficiaient somme toute à peu de monde. Non seulement vous ne faites pas de même pour les niches comme la « niche Copé » qui coûte très cher aux finances publiques, mais vous les élargissez. Ainsi, les plus-values de cession, aujourd'hui taxées à 12 %, le seront demain à 5 % ! Il est à craindre que le renforcement du mécanisme d'exonération d'imposition sur les plus-values de deux ans et plus ne crée un appel d'air pour certains grands groupes qui ont d'ores et déjà recours massivement au dispositif. Or, malheureusement, il a été constaté dans de nombreux cas que le régime d'intégration des groupes est très souvent utilisé comme l'un des principaux outils de l'optimisation fiscale. Quel

l'élargissement de la niche fiscale. Le Gouvernement établit assez clairement que la France dispose d'ores et déjà d'un régime d'intégration fiscale plus favorable que les autres pays européens. la première partie de l'article 12 correspond à une hausse de la fiscalité pour les entreprises concernées afin de nous mettre en conformité avec le droit européen, cela vient d'être indiqué.

afin que la « niche Copé » ne soit pas augmentée. Je partage par ailleurs l'avis de notre collègue Éric Bocquet quant au chiffrage de la réforme de ce régime d'intégration, sur lequel nous ne disposons pas d'éléments suffisamment précis.

la taxation à 12 %, sauf pour les cessions intragroupes, pour lesquelles ils ont conservé le taux de 5 % proposé par le Gouvernement. Comme indiqué par le ministre de l'économie et des finances au cours des débats, la France est le seul pays à taxer à un seul taux. Dans les autres pays européens, ces entreprises sont majoritairement totalement exonérées ou soumises à un taux de 5 % au plus. Le projet initial du Gouvernement permettait d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il convient donc d'y revenir. Quel est l'avis de

Elle peut aussi ne plus remplir les conditions propres à l'option qu'elle a exercée alors qu'elle remplit celles d'une autre forme de groupe fiscal. Actuellement, lorsqu'une société mère substitue une nouvelle option à celle qui était initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d'ensemble les sommes qui n'ont pas été

en additionnant les résultats propres des sociétés membres, déterminés dans les conditions de droit commun. Serait ainsi obtenu le résultat imposable du groupe. Tout en recherchant l'objectif de mise en conformité européenne du régime de groupe fiscal, ce dispositif constitue une grande simplification

qui leur prend beaucoup de temps. Pour ces groupes de PME, le résultat d'ensemble imposable est déjà celui qui correspondrait au cumul des résultats individuels de chacune des sociétés du groupe. Avec ce régime, les groupes ne seraient soumis à aucune opération de rectification ou de neutralisation particulière des opérations intragroupes. Il s'agirait de pratiquer tout simplement la somme algébrique des résultats fiscaux individuels de toutes les entités du groupe pour déterminer le résultat imposable de ce

Merci est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Bocquet. On pourrait s'étonner de voir notre groupe déposer un amendement de suppression d'une directive européenne assez largement inspirée des travaux de l'OCDE sur la lutte contre l'érosion des profits à visée d'optimisation fiscale. savez, tout est dialectique, et il suffit de regarder le véritable concours Lépine de dérogations organisé par les amendements déposés sur le texte de l'article 13 pour se rendre compte que l'affaire n'est pas aussi simple que cela

Quand l'excédent brut d'exploitation d'une entreprise est largement capté par ses actionnaires, quand ce sont des fonds de pension ou des holdings gourmands en rendements à deux chiffres, cela se voit dans le report à nouveau et l'état des fonds propres.

On peut s'étonner tout de même que tant de sollicitude trouve ainsi à s'exprimer à l'endroit de grands groupes dont la surface financière et économique est déjà suffisamment étendue pour savoir jouer des différents ressorts de l'optimisation fiscale. Quel est l'avis de la commission

du court terme et d'une dictature des actionnaires. Les actifs financiers et les actifs liquides et monétaires détenus par les entreprises non financières qui thésaurisent ainsi leur excès d'épargne représentent aujourd'hui environ 175 % du PIB en valeur pour l'ensemble de l'OCDE,

Transposer, oui ; surtransposer, non ! L'article 13 tend à transposer l'article 4 de la directive ATAD, qui vise à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Pour cela, il réforme le régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Il limite notamment à 30 % de l'EBITDA- -la déductibilité par une entreprise non membre d'un groupe. Cette mesure, hélas, impacte

prévoit, certes, que les projets pour lesquels une procédure d'attribution a été lancée avant la promulgation du présent projet de loi de finances seront exemptés du nouveau cadre fiscal, mais il n'est pas certain, en l'état de la rédaction proposée, que les projets d'énergie marine renouvelable concernés seront bien inclus dans le champ des projets visés aux 1° à 5° du 1. du III que vise à ajouter l'amendement. Or l'imposition de nouvelles règles de limitation des charges financières

avec des projets d'infrastructures publiques de long terme- je pense en particulier au soutien public dont ils bénéficient, qui s'exprime au travers d'un contrat de nature administrative -et qu'ils répondent à un objectif d'intérêt général, fixé par la loi. Les sociétés de production d'énergie renouvelable sont par ailleurs, du fait des caractéristiques des installations de production qu'elles mettent en oeuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, avec un recours à la dette généralement à hauteur de 80 %. Par cohérence avec les objectifs de la politique énergétique et pour éviter un renchérissement des projets d'énergies renouvelables, qui serait payé par le contribuable, le présent amendement vise à ajouter à la liste des exceptions les projets d'énergies renouvelables électriques ou gazières, sur terre et en mer, au même titre que les autres projets d'infrastructures publiques de long terme.

Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette, généralement à hauteur de 80 %. L'article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l'article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en oeuvre un nouveau mécanisme d'encadrement de la déductibilité des surcoûts d'emprunt, seront déductibles sous réserve d'un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d'euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières. Le dispositif qui fait l'objet de l'article 13 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables et pénalise ainsi leurs activités, sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire, avec pour objectif la fraude, alors même qu'elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé, de la nature de l'investissement, réalisé intégralement et massivement au début du projet. Pour cette raison, la directive ATAD permet de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l'objet d'une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d'infrastructures publiques de long terme. À cet effet, une liste limitative d'exceptions pour les cocontractants de l'administration a été introduite

Elles occupent en effet une part croissante dans la production d'énergie et présentent des similitudes avec d'autres installations identifiées comme des infrastructures publiques de long terme. Nous souhaitons que les sociétés du secteur des énergies renouvelables ne soient pas pénalisées dans leurs activités. Rappelons que la directive du 12 juillet 2016 permet,

ce qu'ils permettent de satisfaire un besoin collectif. Reconnaissons aussi qu'ils permettent de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés à l'horizon 2030, notamment le taux de 40 % d'électricité renouvelable. J'ajoute que les projets éoliens en mer nécessitent des années d'études, de construction

des titres remis en contrepartie d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité, une BCA, ou d'éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1 janvier 2018, lorsqu'elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions. Le présent amendement prévoit que l'entreprise apporteuse reprenne l'antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l'apport. Cette mesure s'applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d'un apport partiel d'actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il paraît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés, afin que l'opération de restructuration demeure neutre fiscalement.

Il est demandé que les PME qui s'engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d'impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun. Pour améliorer l'attractivité de notre pays et attirer les investissements, il est proposé l'instauration d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les résultats réintégrés au capital des PME patrimoniales. Si l'on veut dynamiser l'investissement en augmentant les capacités de financement des PME, il convient de mettre en place un instrument les incitant à investir. Cette mesure permettrait de soutenir les PME dans leur activité. concernée pourrait alors acquérir davantage de visibilité en matière d'investissement et continuer à renforcer ses fonds propres sans redouter la combinaison d'aléas conjoncturels et d'une taxation impactant sa trésorerie.

Cet amendement vise à ajuster la trajectoire de baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés prévue l'an dernier à l'article 84 de la loi de finances pour 2018 afin d'aligner, à l'issue du quinquennat, le taux français sur le taux moyen européen, soit 23 %. Avec un taux normal d'impôt sur les sociétés abaissé à 25 % à l'issue du quinquennat, et sans tenir compte des baisses à venir dans les autres États européens, la France continuera en effet à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne. À situation inchangée dans les autres États membres de l'Union européenne, dix-neuf d'entre eux auraient encore en 2022 un taux inférieur à celui de 25 %. La France a besoin d'un choc d'attractivité pour en finir avec une croissance atone. Nous ne devons pas craindre une baisse de recettes : l'exemple britannique a montré que les recettes d'impôt sur les sociétés augmentaient à mesure que baissaient les taux. L'économie est un jeu non pas à somme nulle, mais à somme positive. La création de richesses dépend donc, en amont, des incitations qui sont délivrées aux entrepreneurs.

nous devons aussi tenir compte de la structure de nos impôts et du caractère très défavorable des impôts de production, la commission émet un avis défavorable

les dépenses en matière de recherche et développement dans les sociétés privées, notamment d'aider l'emploi des chercheurs au sein de ces sociétés. Le dispositif actuel constitue une aide à l'externalisation de cette recherche dans des organismes publics,

Je ne peux pas accepter votre argumentaire, monsieur le rapporteur général, puisque le taux de 200 % est utilisé par certaines sociétés pour abandonner toute recherche interne et externaliser la totalité de la recherche et développement à l'extérieur, dans des sociétés publiques. De la sorte, on n'encourage pas du tout la mutualisation de la recherche et la collaboration des deux acteurs, auxquelles je suis favorable. Au contraire, on favorise une externalisation absolue. Je

but est de rester compétitifs pour ne pas faire partir nos sociétés vers des pays qui ont fixé un impôt sur les sociétés beaucoup plus bas. Le risque est effectivement que les sociétés quittent le territoire pour aller en Irlande et vers tous les pays que notre collègue Éric Bocquet a cités tout à l'heure.

qui vise à abaisser à 7 % le taux préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets dans le cadre du nouveau régime prévu. Je rappelle que l'Assemblée nationale avait abaissé ce taux à 15

de déroger au principe du « nexus » en appliquant un ratio de remplacement sans perdre le bénéfice du taux réduit relatif aux brevets. Cette procédure a vocation à être exceptionnelle. Elle est très encadrée par l'OCDE. C'est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de la conditionner à l'obtention d'un agrément préalable. Quel est l'avis de la commission ? Favorable. Je mets aux

du projet de loi de finances pour 2019 modifie le champ d'application de l'avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables, mais non brevetées, qui bénéficiaient jusqu'ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets. L'objet du présent amendement est de permettre à l'ensemble des titres de propriété industrielle définis et protégés par le code de la propriété intellectuelle français de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l'OCDE. Par ailleurs, cet aménagement permettra de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du rapport de l'OCDE, s'adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française.

réduit d'impôt sur les sociétés, à 19 %, sur les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2022 sous condition d'un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements. Ce dispositif ne s'applique que dans les zones tendues. loi ÉLAN, comprend plusieurs mesures incitant les organismes d'HLM à se regrouper et à se restructurer, ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Il paraît utile de mettre en place ce taux réduit d'IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux vers la construction de logements locatifs sociaux. Cet amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant l'application du taux de 19 % aux plus-values immobilières réalisées par les organismes d'HLM à l'occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

général des impôts dispose qu'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficie d'une taxation à taux réduit de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements. Ce dispositif est utilisé, en particulier, pour faire muter des espaces logistiques, des ensembles de bureaux, des entrepôts, dans le tissu urbain dense. L'article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2020, mais il en a aussi resserré le champ d'application, en le réservant aux zones A et

en vigueur pendant une quinzaine d'années pour alléger l'ISF, dont il ne vous aura pas échappé que nombre de nos concitoyens réclament aujourd'hui le rétablissement. Ce dispositif des engagements collectifs de conservation entendait répondre aux problèmes posés par la situation des actionnaires minoritaires dépourvus de fonction dirigeante au sein des entreprises et groupes dont ils détenaient des parts. L'article 16 prévoit d'assouplir les conditions d'exercice des droits associés à ces pactes et s'apparente, à bien y regarder, à une sorte d'extension de la loi sur le « droit à l'erreur » dont nous avons débattu voilà quelques mois ici même. le texte revient à parer à toute éventualité pour assurer autant que faire se peut la conservation du patrimoine que constitue l'entreprise : il s'agit d'étendre le bénéfice du « dispositif Dutreil » en abaissant les seuils de détention. La valeur d'une entreprise doit beaucoup- chacun le sait -, bien sûr, non seulement à l'imagination et à la créativité de ses dirigeants, mais aussi au travail de ses salariés. La perception de droits de mutation en cas de transmission n'est, d'une certaine manière, qu'un juste retour des choses : une contrepartie de la valeur créée par le travail de la collectivité.

aux entreprises individuelles

un assouplissement utile.

entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l'objet de l'engagement collectif de conservation. Ce nombre maximal de niveaux d'interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes industriels familiaux, dans lesquels, au fur et à mesure que des transmissions successives se produisent, le capital se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus nombreuses. Une nouvelle transmission qui intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire ces derniers à souhaiter constituer leur propre holding. En outre, compte tenu du mécanisme de prorata prévu par le b de l'article 787 B du CGI, seule la fraction de la valeur des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue dans la société industrielle peut bénéficier de l'exonération, mais non pas les autres actifs pouvant éventuellement être détenus par la holding : cet article prévoit déjà qu'en présence de plusieurs degrés d'interposition ce prorata est appliqué à chaque niveau, empêchant tout effet d'optimisation. Si admettre un plus grand nombre de niveaux d'interposition n'entraîne donc aucun risque de disparition d'assiette imposable, le contrôle fiscal s'en trouve néanmoins compliqué. C'est pourquoi cet amendement tend à porter à trois le nombre maximum de niveaux d'interposition entre le redevable et la société

du Gouvernement ? Tout l'objet de l'article 16 est de permettre les transmissions et de favoriser la préservation du capital sur le sol français. Nous considérons toutefois que le bénéfice du pacte Dutreil constitue un avantage fiscal particulièrement dérogatoire, qui fait déjà l'objet d'assouplissements ; il ne convient pas de l'assouplir davantage, au risque de rendre cet avantage disproportionné. Par ailleurs, l'exonération partielle est intrinsèquement liée à la nécessaire et forte implication du redevable dans l'entreprise. Il nous semble qu'ajouter un troisième niveau d'interposition risque en réalité de distendre le lien entre l'actionnaire initial

de holding pour permettre l'arrivée d'actionnaires nouveaux sans priver la famille du contrôle. Certes, ces systèmes de poulies peuvent surprendre ; mais c'est là le prix à payer pour combattre cette particularité très républicaine inhérente au droit français, celle de la division du patrimoine à chaque génération. La seule façon de lutter contre cette division est de faire venir des actionnaires nouveaux en acceptant qu'ils soient minoritaires. Cela fait des étages en plus, et le bonheur des avocats ; mais il y va de la transmission des entreprises et de leur continuité.

pouvoir bénéficier du pacte Dutreil, d'exercer les fonctions de direction pendant la phase d'engagement collectif et pendant une durée de trois ans à compter de la transmission. Si le dirigeant

de conservation lorsque leur détenteur accepte l'échange de ses titres dans le cadre d'une offre publique préalable à une fusion ou à une scission. Cependant, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l'engagement souscrit par le redevable auteur de l'échange soit contraint d'abandonner ses fonctions. Cela peut se produire chaque fois que les associés de l'entité qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la restructuration ont la capacité et décident effectivement de l'évincer. Cet amendement tend donc à délier les bénéficiaires de la transmission de l'exigence posée par le d de l'article 787 dans des circonstances de fusion, de scission ou d'offre publique d'échange. Cet assouplissement est de nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises : celles-ci doivent pouvoir fusionner ou se scinder sans devoir obligatoirement maintenir jusqu'au bout le dirigeant ayant souscrit l'engagement initial de conservation des titres.

du Gouvernement ? Il nous paraît assez logique que, lorsque les actionnaires d'une entreprise liés par un pacte Dutreil cèdent l'entreprise et leurs participations, ce pacte tombe.

vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial, dès lors que les titres sont conservés pour une durée de dix ans. Cette mesure s'inspire d'une proposition formulée par notre excellent collègue Olivier Cadic

Si nous voulons « muscler » l'appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises, nous devons prendre une mesure forte, à savoir l'exonération totale de droits de mutation, comme en Suisse, en Russie, au Portugal ou au Royaume-Uni.

Des risques constitutionnels existent, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques ; nous ne les ignorons pas. C'est la raison pour laquelle nous proposons de subordonner le bénéfice de l'exonération à l'engagement de conserver les parts de l'entreprise pour une durée de dix ans, au lieu de six ans aujourd'hui. En outre, comme l'a souligné Olivier Cadic dans son rapport, un motif d'intérêt général justifie ici une exonération fiscale exceptionnelle : l'intérêt national est mentionné dans un commentaire autorisé d'une décision constitutionnelle relative aux droits de succession.

présenterait un caractère central mais pas exclusif. En particulier, il reviendrait à la doctrine administrative, à l'issue de négociations avec les professionnels, de prévoir des mesures de tolérance lorsque les autres actifs détenus par la holding sont intimement liés à l'activité opérationnelle des filiales.

Or, à ce jour, l'augmentation de ce taux n'a pas été validée par la Commission européenne. Les investisseurs ne savent donc toujours pas quelle réduction d'impôt leur sera applicable, ce qui crée un attentisme, au rebours de l'intention sous-tendant la mesure voulue par la majorité.

ce qui incite de nombreux dirigeants à suivre des stratégies d'optimisation fiscale reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise. Ce processus s'avère bien souvent plus coûteux que prévu et constitue un effet pervers auquel le présent amendement vise à mettre fin

Le présent amendement a pour objet d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, sous réserve d'un engagement à les conserver cinq années supplémentaires au au terme de la durée de conservation visée au premier alinéa de l'article 793 du code général des impôts portant sur les mutations à titre gratuit. L'exonération de 75 % s'applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq ans ; en deçà de cette limite l'exonération est ramenée à 50 %.

fait, les successions familiales sont de moins en moins nombreuses, et les ventes à la découpe se multiplient. Les conséquences en sont lourdes pour le tourisme français, qui doit faire face à une forte concurrence internationale.

Cet amendement, dont mon collègue Raymond Vall est le premier signataire, a déjà été présenté lors de l'examen de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise. Notre objectif est de répondre aux risques financiers auxquels peuvent être exposés les héritiers d'une entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant.

à terme, dans la mesure où la valorisation de l'entreprise peut évoluer fortement, y compris à la baisse, sans indexation des droits à payer. Conformément à l'ambition du Gouvernement et dans la perspective du projet de loi PACTE, il est dans l'intérêt du pays, des entreprises et des territoires de rechercher des solutions à cette question.

Le référé 2017-1860 précisait d'ailleurs que le Gouvernement devait engager une réflexion sur les modalités de mise en oeuvre de l'imposition, qui passerait par la création de mécanismes permettant d'assurer la territorialité de l'impôt et par une redéfinition du fait générateur, la livraison d'un titre s'effectuant non le jour de la transaction, mais deux jours plus

aux transactions intrajournalières. Dites, ces transactions interviennent avant le transfert de propriété à l'acquéreur et sont dénouées au cours d'une seule et même journée. journée. Elles incluent notamment les transactions à haute fréquence, consistant à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers, grâce à des programmes informatiques Les transactions à haute fréquence représentent, selon l'autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris. Cet amendement vise deux objectifs d'une part, dégager des recettes fiscales supplémentaires, en vue notamment d'augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques ; d'autre part,

objectif est d'augmenter les recettes fiscales liées aux transactions financières, afin d'accroître la participation du secteur financier aux recettes de l'État. En 2018, 142 entreprises sont concernées, le montant de leur capitalisation boursière étant supérieur à 1 milliard

et le paludisme, un engagement fort de notre pays dans l'aide publique au développement, avec un rebond capable de constituer un véritable marqueur, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, aurait été bienvenu. Dans ce cadre, l'augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières constituerait un message à la hauteur des enjeux et permettrait de rappeler la vocation même de la TTF, à savoir faire participer la finance et les acteurs spéculatifs au développement, eu égard à l'ensemble des investissements publics dont ils bénéficient et à leur implication dans le creusement des inégalités constaté de rapport en rapport chaque année.

pour financer la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques. Selon de nombreuses associations- Oxfam, Coalition PLUS, etc. -, l'augmentation du taux de la TTF

à M. Éric Bocquet. L'article 150 U du code général des impôts exonère les particuliers de l'impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'organismes chargés du logement social jusqu'au 31 décembre 2020. 31 décembre 2020. Nous proposons d'élargir la liste des organismes de logement social visés à deux nouveaux types de structures. Je rappelle que cette liste comprend aujourd'hui les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, l'association Foncière Logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, ainsi que les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage. Il est proposé que l'exonération s'applique également en cas de cession à une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes d'HLM détiennent la majorité des parts. En effet, ces organismes constituent parfois, pour les besoins de leurs opérations de réalisation de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » ces opérations. En application du code de la construction et de l'habitation, l'objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes d'HLM qui les ont constituées,

Je rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d'acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires au titre de la location ou de l'accession à la propriété des logements à usage d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyer et de prix de cession.

le CGI, exonère les particuliers de l'impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'organismes chargés du logement social jusqu'au 31 décembre 2020.

Le ministre du logement a indiqué il y a quelques jours à Lille que le dispositif des OFS « est une des solutions qu'il faut absolument développer pour permettre le logement abordable ». Pour démultiplier ce dispositif, nous proposons une mesure d'incitation fiscale.

ce régime d'abattement ne s'applique que dans les zones tendues, et uniquement à condition que l'acquéreur du terrain s'engage à construire dans les quatre ans des logements neufs. Or un OFS ne peut pas prendre un tel engagement, dès lors que c'est non pas lui qui va construire, mais un autre opérateur. En outre, les opérations de bail réel solidaire ne portent pas toujours sur des constructions neuves ; elles peuvent également concerner des logements anciens.

aussi les cessions réalisées au profit de SCI dont les parts sont majoritairement détenues par des organismes chargés du logement social.

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements. Il est proposé d'étendre l'exonération prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts en faveur du logement social aux cessions réalisées au profit de sociétés civiles immobilières détenues majoritairement par des organismes d'HLM ou des organismes de foncier solidaire. Si les SCI visées par l'amendement

disposent d'un revenu moyen d'environ 190 000 euros. Concernant la réforme de la taxe d'habitation, les choses sont plus simples : l'État est censé avoir perdu environ 1,3 milliard d'euros en 2018 et devrait perdre quelque 1,9 milliard d'euros les années suivantes. Nous ne savons pas quel est l'effet exact du PFU sur le produit de l'impôt sur le revenu, mais on évoque tout de même une nouvelle perte de 330 millions d'euros cette année. Si l'on rapproche les sommes indiquées du nombre de contribuables potentiellement bénéficiaires de la mesure,

Le traitement fiscal différencié entre capital mobilier et capital immobilier repose sur le postulat erroné suivant lequel les actifs immobiliers ne seraient pas productifs.

Ce système de, traitant distinctement revenus du travail et revenus du capital, mais avec un taux de l'impôt frappant les revenus du capital uniforme et relativement faible, existe dans plusieurs pays nordiques depuis le début des années

pèsent tout de même, je vous le rappelle, mes chers collègues, 17 % de la valeur ajoutée française, ne seraient pas productives. La politique du Gouvernement, avec le remplacement de l'ISF par l'IFI, la réforme de la taxe d'habitation, va immanquablement aboutir à un transfert massif de l'imposition vers le foncier bâti, alors même que la France est le pays d'Europe où la propriété immobilière est déjà le plus fortement taxée.

immobilière. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader l'investissement privé dans l'immobilier. Je suggère que nous adoptions cet amendement, qui ne règle pas tout, tant s'en faut, mais qui a l'immense mérite de poser le problème et d'obliger le Gouvernement à faire mouvement sur ce sujet extrêmement sensible.

est ainsi libellé : La parole est à M. Fabien Gay. À notre sens, la fiscalité du patrimoine appelle un certain nombre d'évolutions. De fait, nous proposons d'appliquer à la capitalisation de l'assurance-vie le traitement que l'on réserve, pour l'heure, aux successions et donations de biens.

dispositif. Pour l'heure, sont éligibles l'ensemble des « organismes reconnus d'utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d'assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l'environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture,

Il n'est pas nécessaire de le gager, puisque, d'après les estimations disponibles, son adoption permettrait d'accroître les recettes fiscales de l'État d'environ 4,7 milliards d'euros.

estiment que cet effort doit être mieux réparti. Il n'est pas acceptable de fragiliser les catégories de population modestes,

! Les auteurs du présent amendement estiment qu'une répartition plus équitable de l'effort fiscal, en fonction des moyens contributifs de chacune et de chacun, est plus propre à relancer la croissance par la consommation, plus efficace en termes de lutte contre les inégalités et plus légitime sur un plan philosophique. Mes chers collègues, aucun argument sérieux ne permet de légitimer le maintien de ce dispositif, qui renforce les inégalités et ressemble de plus en plus au bouclier fiscal de sinistre mémoire. Quand le temps des illusions laisse la place au temps des soustractions, il faut savoir parler aux Français, monsieur le secrétaire

c'est de mettre un terme à certains dispositifs inégalitaires. La réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune et autres mesures en faveur des catégories aisées font partie de ces dispositifs inégalitaires aujourd'hui massivement rejetés. Comment accepter, en effet, que le sommet de la pyramide bénéficie d'un allégement d'impôt de quelque 5 milliards d'euros, tandis qu'un très fort pourcentage de Français

répartir plus équitablement l'effort demandé, contribuerait à réduire les inégalités et donnerait au Gouvernement quelques moyens supplémentaires pour compenser

des valeurs qui, sans aucun doute, pèseront bien plus lourd que le prétendu ruissellement ! La parole

de Londres le 21 février 2017 : « Dans mon programme, vous aurez une série d'initiatives pour attirer les gens de talent dans la recherche, et dans de nombreux autres domaines. [ ...] Je veux les banques, les talents, les chercheurs, Cela fera partie de mon programme de les attirer. [ ...] Je veux les convaincre que la France change [ ...], qu'ils auront l'opportunité de revenir en France dans les prochaines années et d'y rencontrer le succès. » La suppression de

Londres, peut-être quelques centaines en Belgique et en Suisse : ceux-là ont fait leur vie. Ce que je souhaite, c'est que ceux qui ont leur vie à faire la fassent en France, qu'ils aient confiance dans la capacité de notre pays à respecter durablement le fruit de leur travail

combien ont échoué ? Il faut reconnaitre le droit au succès, comme il faut d'ailleurs admettre le droit à l'erreur. Sans cela, il n'y aura pas d'économie vivante. Les millions de salariés qui ont besoin d'entrepreneurs,

même niveau ! Mes chers collègues, nous vivons une période difficile, dangereuse, où l'essence même de notre démocratie peut être remise en cause.

des recettes fiscales supplémentaires qui seraient bien utiles dans la période que nous connaissons et permettraient au Gouvernement de répondre à la demande formulée par toutes ces personnes qui manifestent. Au-delà,

des organismes internationaux que l'on ne pourra pas taxer de gauchisme, comme l'OCDE ou le Fonds monétaire international, soulignent que que la question des inégalités est un sujet majeur, dont le traitement conditionne le devenir de nos sociétés.

les sociétés les plus dynamiques, y compris en termes de création de richesses, sont celles qui sont le moins inégalitaires.

totalement irrationnelle le prix du foncier agricole. Je peux vous parler du Médoc, de Pomerol, de la Gironde ; mes collègues vous parleront de la Champagne ou de la Bourgogne. Les prix à l'hectare grimpent en flèche et l'on assiste dans le même temps à une concentration des exploitations. de ce constat, j'avais proposé l'an dernier un dispositif visant à favoriser la transmission familiale et à préserver notre modèle agricole français. Vous l'aviez écarté, au motif qu'il fallait attendre la loi de finances de 2019 pour introduire une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole. préventif, j'ai poursuivi ce travail et j'ai remis à Bruno Le Maire, voilà quelques semaines à Bordeaux, une proposition de loi cosignée par une cinquantaine de collègues sénateurs. Le présent amendement est issu de ce travail collectif.

Aujourd'hui, l'IFI pénalise les paysans et les vignerons. L'exemple des propriétaires historiques de l'île de Ré déracinés par la flambée des prix doit vous servir de leçon. servir de leçon. Mes chers collègues, je vous demande un soutien plein et entier à cet amendement, afin d'envoyer un signal positif à nos viticulteurs en cette période tourmentée.

a opportunément permis d'exonérer les actifs financiers. Cette réforme a constitué un premier pas, certes utile, mais insuffisant. L'IFI reste une énième exception française, au détriment de l'attractivité de notre pays et de ses investissements productifs. L'harmonisation fiscale européenne, que j'appelle de mes voeux, n'a aucune chance d'aboutir si elle n'est invoquée que pour masquer les défauts les plus criants de notre système fiscal et l'indiscipline de nos politiques budgétaires.

Le Gouvernement affiche la sauvegarde du patrimoine culturel bâti comme l'une de ses priorités. Il en parle beaucoup, on l'aura remarqué ... Pourtant, 7 % des 44 000 bâtiments classés monuments historiques en France, dont une part importante est aux mains de propriétaires privés, sont en situation de péril.

ne peut pas être considérée comme une source de rente. À ce titre, elle ne répond pas à la logique qui a présidé à la création de l'IFI, à savoir réorienter le patrimoine immobilier vers le financement de notre économie. Nul ne vendra jamais sa résidence principale pour investir dans l'économie réelle ! En outre, les propriétaires ne peuvent pas être tenus pour responsables des évolutions du marché immobilier, qui peuvent être telles que certains propriétaires, pourtant non redevables de l'impôt sur le revenu, se retrouvent assujettis à l'IFI. Cet amendement vise à porter la déductibilité de la valeur de la résidence principale à un niveau susceptible de mieux

Le dispositif de l'intermédiation locative constitue l'une des réponses au problème de la vacance : il permet de mobiliser des logements privés et de les prendre à bail pour loger des personnes aux revenus modestes. Le principe en est simple : une association est locataire d'un logement privé qu'elle sous-loue à une personne contre un loyer compatible avec les moyens de celle-ci, tout en en assurant l'accompagnement social. Ainsi, le propriétaire est garanti tant contre les impayés une garantie financière que contre les difficultés de tous types et les dégradations- il s'agit des deux freins psychologiques à la location d'un logement à une personne aux ressources faibles. L'objectif est d'inciter les personnes physiques concernées par l'IFI à mettre en location leurs biens immobiliers dans le cadre de dispositifs solidaires et de favoriser ainsi la location

immobilière, soit une diminution de 16 % sur un an. La collecte réalisée auprès des particuliers en 2017 avait permis de recueillir 21 millions d'euros au total. Ce recul de la collecte auprès des particuliers fortunés doit être replacé dans le contexte d'une baisse générale de la collecte auprès du grand public en raison de la hausse de la CSG, qui touche notamment les retraités, donateurs traditionnels, et des incertitudes liées à la mise en oeuvre du prélèvement à la source à partir de 2019. Afin de compenser partiellement la perte de ressources consécutive au passage de l'impôt sur la fortune à l'impôt sur la fortune immobilière et de conserver les grands donateurs, il est proposé d'instaurer une mesure fiscale visant à inciter les particuliers assujettis à l'IFI à effectuer un don plus important.

La transformation de l'ISF en IFI a eu pour effet de faire baisser le nombre des redevables de 350 000 à 136 000.